La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 prises pour son application, la commission des lois s'est prononcée, lors de sa réunion de ce jour, par 7 voix pour et 7 voix contre, sur le projet de nomination de Mme Dominique Simonnot aux fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

un rappel au règlement portant sur la place du Parlement en général, et de la Haute Assemblée en particulier, dans le débat qui nous attend sur la prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet dernier.

Quelles que soient les urgences, monsieur le ministre, le respect du Parlement doit être une préoccupation permanente de notre gouvernement et de l'exécutif, en particulier du Président de la République.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

Ce n'est pas la première fois que je me trouve devant vous pour examiner un texte ayant trait, de près ou de loin, à l'état d'urgence sanitaire. Lorsque nous nous étions vus pour la dernière fois, nous avions débattu de la durée

monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est la quatrième fois que nous sommes amenés à légiférer sur les pouvoirs que nous consentons au au Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Il y a eu successivement deux régimes, l'un d'état d'urgence sanitaire, l'autre qualifié de « sortie » de l'état d'urgence sanitaire. Mais c'est une sortie qui n'en finit pas, puisque le Gouvernement nous demande maintenant de prolonger ladite sortie jusqu'au mois d'avril 2021. Autant dire que ce texte est déjà mal nommé : c'est en réalité un texte de prolongation des pouvoirs exceptionnels que le Gouvernement estime nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire, qui rebondit actuellement. La seule différence entre le régime de l'état d'urgence sanitaire et le régime dit de « sortie de l'état d'urgence sanitaire, c'est que, dans la deuxième hypothèse, le Gouvernement n'a pas le droit de prononcer le confinement généralisé de la population tel que nous l'avons connu du mois de mars au mois de mai. Encore Encore faut-il se rappeler que la loi de mars dernier sur l'état d'urgence sanitaire reste en vigueur, et que le Gouvernement peut à tout moment par décret déclencher le régime du confinement généralisé. Évidemment, c'est l'instrument de dernier recours, et nous ne blâmons pas le Gouvernement de ne pas s'inscrire dans cette perspective, qui ne pourrait être acceptée que dans une situation de crise tellement grave qu'il faudrait de nouveau interrompre l'activité nationale. Notre espoir, depuis la fin du confinement, est au contraire de réussir à lutter contre l'épidémie sans avoir à suspendre l'activité économique et sociale de notre pays. C'est sans doute une mais nous mesurons à quel point le confinement généralisé est la mesure à laquelle il a fallu recourir faute de mieux, et à défaut d'avoir été préparés à affronter une telle épidémie. Il est vrai que, au mois de mars dernier, nous n'avions pas de masques, pas de gel hydroalcoolique, pas de tests de dépistage accessibles à la population et, surtout, pas de système national d'information permettant de remonter les filières de contamination en neutralisant les personnes exposées à la contamination le temps que l'on vérifie leur statut au regard de l'épidémie. Au fond, la sortie de l'état d'urgence sanitaire se réduit à un enjeu faire en sorte que l'on substitue de multiples confinements individualisés et temporaires au confinement généralisé de la population.

de personnes qui ont pu être diagnostiquées comme porteuses du virus grâce au système national d'information mis en place et aux plateformes de l'assurance maladie, qui ont recherché ce qu'il est convenu d'appeler les cas contacts. La situation actuelle, qui préoccupe tous les Français, et particulièrement nos autorités sanitaires, est une situation de très nette aggravation

que celle que nous avons connue au mois de mars dernier, elle est cependant suffisamment préoccupante pour qu'il n'y ait pas à débattre de l'opportunité de prolonger les pouvoirs exceptionnels que nous avons accordés au Gouvernement au fil des lois que nous avons débattues ici même. Nous avons donc admis, à la commission des lois, le principe la poursuite de cette action qui restreint l'exercice des libertés individuelles et des libertés publiques pour réduire les risques de contamination. Nous attendons, bien sûr,

c'est-à-dire au-delà du 31 janvier prochain. J'ai bien entendu votre argument, mais je dois vous dire que nous ne souhaitons pas non plus vous laisser mettre en place le système permanent de pouvoirs exceptionnels par la loi que vous voulez nous faire adopter, et dont nous ne savons rien à ce stade. Il est donc très difficile pour nous de vous donner une sorte de blanc-seing, en vous laissant appliquer ces pouvoirs exceptionnels, non pas pendant deux ou trois mois, comme ce fut le cas avec les précédentes lois, mais pendant une très longue durée, au seul motif que vous avez l'intention de nous faire adopter un régime permanent de pouvoirs exceptionnels pour restreindre les libertés en vue de lutter contre cette épidémie ou de nouvelles à venir. Nous sommes donc très fermes sur cette exigence du contrôle parlementaire. Il s'agit tout de même de choses essentielles pour la vie des Français, et je crois que notre vocation, en tant que représentants de la Nation, est bien de consentir au Gouvernement les moyens nécessaires à l'efficacité de la lutte contre l'épidémie, mais d'exiger aussi en retour que nous puissions assumer notre responsabilité de contrôle dans sa plénitude. Je voudrais vous dire par ailleurs, monsieur le ministre, que nous souhaitons apporter notre contribution, comme nous l'avions fait au mois de juillet, à votre volonté de réformer les régimes de lutte contre les épidémies, en mettant à jour ce fameux article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui aujourd'hui

Si cet article avait été appliqué sans que l'on adopte la loi relative à l'état d'urgence sanitaire, vous auriez eu de très graves difficultés juridiques. C'est bien la preuve qu'il n'est pas adapté à ce genre de situations. Nous voulons donc le modifier. Enfin, nous avons pris un certain nombre de mesures, qui nous ont été inspirées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), pour ce qui concerne les fichiers utilisés pour lutter contre les risques de contamination ou procéder à des recherches épidémiologiques. Nous avons également souhaité que des dispositions soient prises pour préparer les scrutins de mars 2021. La démocratie est une affaire trop sérieuse pour

le vote par correspondance, en lui apportant des garanties qui lui ont fait défaut dans le passé- raison pour laquelle il avait été supprimé de notre code électoral ? La commission des lois, dans une forme d'unanimité, a souhaité

afin que le scrutin de mars prochain se déroule dans de bonnes conditions, quelle que soit l'intensité de l'épidémie à cette date. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà ce que je tenais à vous dire au moment d'ouvrir ce débat. L'heure est manifestement grave. Le Sénat est au rendez-vous, mais ne consentira pas à accorder des pouvoirs dérogatoires au Gouvernement sans de sérieuses garanties.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, 32 683, il s'agit là d'un sinistre nombre, celui des morts du covid-19 en France. Force est de constater que davantage aurait pu être fait par l'exécutif, non pas au coeur de la crise, quand le Gouvernement s'est finalement résolu à aligner les milliards d'euros, mais bien en amont. Le sous-investissement dans le système hospitalier français n'est pas nouveau : coups de rabot dans les budgets, privatisation totale ou partielle de certains établissements. Les gouvernements successifs de ces dernières décennies se gardent bien de reconnaître leurs erreurs en matière sanitaire et sociale. Le constat est pourtant implacable : les politiques menées

Ne pensez-vous pas que ces places auraient pu être utiles en avril, alors que nos médecins étaient surchargés face aux vagues de contamination ? Cela fait des années que, dans ma circonscription parisienne, les services de réanimation se trouvent saturés et que des patients se voient réorientés vers Chartres ou Orléans. Pour quelles conséquences ? Des patients moins bien soignés qu'auparavant, ainsi que des médecins qui, découragés par ces conditions de travail iniques, abandonnent l'hôpital pour la recherche ou le privé. C'est tout notre système de santé qui est en déliquescence, et le modeste Ségur de la santé n'est pas de nature à nous rassurer. En mars, la réponse du Gouvernement à l'épidémie a d'abord été l'état d'urgence sanitaire et le confinement. Bien que contraignant, ce dispositif a sans aucun doute été salutaire et aura permis, un temps, de ralentir la circulation du virus. En juillet, l'exécutif a pris la décision de sortir progressivement de l'état d'urgence, mais n'a pas jugé souhaitable de retourner immédiatement au droit commun.

Ce sont ces mesures provisoires que la majorité présidentielle souhaite aujourd'hui proroger de quelques mois : fermeture administrative d'établissements recevant du public, régulation de la circulation des citoyens, encadrement de l'accès aux transports publics pour les usagers, limitation du droit à se rassembler et manifester, création de fichiers informatiques comprenant nombre de données personnelles des malades du covid-19 et de leurs cas contacts afin de retracer les chaînes de contamination. Faisant fi des libertés publiques et individuelles, les droits excessifs confiés au Premier ministre, aux préfets ainsi qu'aux administrations n'ont que trop duré. Mes chers collègues, entre l'état d'urgence sanitaire et le droit commun, il faut choisir. Des mesures transitoires ne sauraient être pérennisées, comme tente aujourd'hui de le faire le Gouvernement. Nous saluons évidemment le travail de la commission des lois et du rapporteur, M. Bas, qui a permis de réduire le délai de prorogation de sortie de l'état d'urgence de deux mois. Mais c'est le principe même de cette prolongation que nous rejetons. Si l'exécutif estime que la situation sanitaire est trop grave pour que le droit commun soit efficace, qu'il prenne la responsabilité d'enclencher l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, permettant la mise en application par décret ministériel de l'état d'urgence sanitaire. L'arbitraire et l'exception ne pouvant devenir la règle, le groupe Écologiste - Solidarité

Ce quatrième rendez-vous était une nécessité, dès lors que le régime transitoire institué par la loi du 9 juillet 2020 arrive à échéance le 30 octobre. Comme l'ont souligné le conseil scientifique et le Conseil d'État lui-même, le retour au droit commun n'est en effet pas de nature à endiguer la reprise, malheureusement bien réelle, de l'épidémie. Cet état de fait sanitaire, qui sollicite notre pleine vigilance- je ne vous apprends rien ! -, s'illustre par les 74 départements en situation de vulnérabilité élevée, les 1 500 personnes atteintes par le covid-19 aujourd'hui prises en charge par les services de réanimation, ou encore l'occupation à hauteur de 40 % des lits de réanimation par des patients en Île-de-France, un taux en progression. d'ailleurs nous alerter sur l'effet d'éviction au détriment de personnes requérant des soins lourds qu'il n'est pas possible de différer de nouveau. Les travaux de contrôle de notre Haute Assemblée ont bien montré la dimension profondément éthique de l'urgence sanitaire.

Le constat ne saurait en lui-même permettre de préjuger avec une évidence certaine du choix du régime juridique adéquat. Là est bien le sujet qui a animé les navettes et les débats successifs dans cet hémicycle. Je salue, à ce titre, la position sur le présent texte de notre rapporteur, qui, suivi par la majorité de la commission des lois, n'a pas remis en cause le principe d'une prorogation du régime transitoire, instituée par la loi du 9 juillet dernier, et qui n'en a pas non plus modifié les contours. Ces derniers avaient d'ailleurs été consolidés par le Sénat lui-même, je veux le rappeler, lors de l'examen en première lecture de la loi du 9 juillet 2020. Les prérogatives conférées au Premier ministre et aux préfets par ce régime ont accompagné une reprise de l'activité et permis une adaptation territoriale de la gestion des résurgences de l'épidémie, ce par une agilité indispensable, comme peuvent en témoigner les modifications successives de l'annexe du décret du 10 juillet 2020 listant les zones de circulation active du virus. L'assise du régime a, en outre, été confortée par la décision de conformité du Conseil constitutionnel, qui a bien précisé que, au terme de nos travaux parlementaires, la faculté d'interdire la circulation des personnes ne pouvait conduire à une interdiction de sortie du domicile. Notre rapporteur s'est également accordé sur les dispositions introduites à l'Assemblée nationale, tout à fait bienvenues, permettant d'adapter le fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales à la situation sanitaire. La commission a enfin utilement confirmé le principe d'une prorogation des systèmes d'information mis en oeuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19 et, par là même, de la conservation des données pseudonymisées aux seules fins de suivi épidémiologique et de recherche sur le virus. Ces systèmes apparaissent en effet indispensables à la mise en oeuvre du triptyque stratégique « tester, tracer, isoler ». Sur ce point, je salue le travail du rapporteur, qui a apporté des garanties juridiques supplémentaires, en tirant notamment les conséquences d'une censure et d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, que le Gouvernement propose de préciser. Finalement, et notre groupe avait déjà pu le dire pour défendre le régime transitoire sous le précédent projet de loi, ce régime pourrait être comparé à la figure mythologique de Janus, non pour le caractère double de son visage qui traduirait ici un faux-semblant ou un état d'urgence déguisé, comme certains persistent à le penser sur ces travées, mais bien au contraire et parce que cette figure incarne la transition entre deux temps, parce qu'elle est orientée vers l'avenir tout en ne se détournant pas du passé, une approche que nous force à adopter la crise sanitaire. Ce soir, c'est précisément sur cette question de temporalité, mes chers collègues, que les positions divergent. La commission a en effet ramené au 31 janvier 2021 l'échéance de la prorogation du régime transitoire et des autres dispositions précitées, que le Gouvernement avait fixée au 1 avril 2021 dans le texte initial. Cette seconde échéance, qui diffère de deux mois de la date de la commission, nous paraît plus opportune et raisonnable en ce qu'elle correspond à l'échéance de l'applicabilité du régime de l'état d'urgence sanitaire, qu'un projet de loi justement présenté en janvier 2021 viendra réviser. Cet alignement n'est pas une position doctrinale. Comme le souligne l'avis du Conseil d'État lui-même, il s'agit de laisser à la disposition du Gouvernement jusqu'au 21 avril une gamme d'outils de réaction à l'évolution de l'épidémie, et de lui permettre d'apprécier, à la lumière d'une à la lumière d'une analyse globale, le régime juridique qui pourrait utilement s'appliquer aux situations de crise sanitaire pour mieux fonder son projet de loi. Dans cette même logique, il semble cohérent de réserver la révision nécessaire de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique à cette réforme plus globale. En conclusion, mes chers collègues, je dirai que des débats importants vont se poursuivre ce soir dans l'hémicycle. Je pense à la durée de prorogation, mais aussi aux mesures visant les adaptations utiles en matière de droit électoral. Je pense enfin aux mesures visant à protéger, s'agissant des loyers, les entreprises faisant l'objet de restrictions dans leur activité professionnelle, ou encore aux mesures visant à adapter les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants de personnes morales, telles que les fédérations sportives.

nous sommes réunis aujourd'hui car la situation de notre pays va nous contraindre, une nouvelle fois, à prolonger un état de fait, ce que je regrette profondément. À la veille de l'allocution du Président de la République, nous pouvons craindre que de nouvelles annonces ne viennent renforcer un état d'urgence qui ne dit pas son nom. La situation que nous connaissons depuis mars est sans commune mesure et nous marquera tous durablement. J'ai, à ce titre, une pensée sincère pour tous nos concitoyens qui sont les premières victimes des mesures, pourtant nécessaires, que nous prenons. Nombreux sont les Français qui ont souffert et qui souffrent encore, soit du covid-19, soit des mesures de restriction de libertés auxquelles la situation sanitaire nous oblige à consentir. Depuis le mois de mars, ces mesures ont un impact sur tous les secteurs économiques de notre pays, qu'il s'agisse de l'artisanat, du commerce, du tourisme, de l'aéronautique, et de bien d'autres secteurs. La vie sociale avec nos proches, les pratiques sportives et culturelles, les sorties au théâtre, au concert, au spectacle, les sorties entre amis, les repas au restaurant sont aussi lourdement impactés.

J'aimerais saluer le courage et la ténacité d'une majorité silencieuse de Français qui respectent les gestes barrières et les règles d'éloignement, bien que ceux-ci suscitent de la frustration et de l'incompréhension. Cette incompréhension et la perte de confiance qui en découle naissent de trop nombreuses volte-face, de retours en arrière, de mesures incompréhensibles de la part du Gouvernement, et de règles parfois difficilement applicables sur le terrain, tout cela à grand renfort de spots télévisuels anxiogènes et d'une communication frénétique. L'augmentation à la fin de l'été de la propagation du virus, du nombre de cas confirmés et d'hospitalisations appelle toutefois notre vigilance. Ces indicateurs épidémiologiques ne sont bien entendu pas les mêmes partout. Car, vous le savez, le virus ne circule pas de manière uniforme sur le territoire. Nous ne sommes certes pas dans la même situation qu'en mars, mais la prudence s'impose si l'on souhaite lutter efficacement contre ce qui s'apparente de plus en plus à une deuxième vague. Pour en revenir au texte, je salue le travail effectué par la commission des lois tout juste renouvelée et par son rapporteur, Philippe Bas. Le raccourcissement à trois mois, au lieu de cinq, de la durée de prorogation du régime de sortie d'état d'urgence sanitaire est une bonne chose, même si lors de nos précédents débats, le groupe RDSE avait regretté que l'on fasse du droit d'exception le droit commun. Force est de constater que nous ne sommes plus réellement en état d'urgence, du fait de la sortie du confinement généralisé, mais que nous sortons du champ du droit commun au vu des dispositions que nous prorogeons aujourd'hui et qui deviennent de moins en moins exceptionnelles. concerne les dispositions prévues aux articles 2 et suivants, les membres de mon groupe et moi-même nous retrouvons dans les mesures ajoutées par la commission, qui apportent certaines garanties en matière d'encadrement de la mise en oeuvre des systèmes d'information. Nous demandions depuis le départ la pseudonymisation de certaines données traitées. Je me félicite de ce qu'elle ait été ajoutée et que la commission se soit rangée à la décision rendue par le Conseil constitutionnel en mai dernier. Autre apport que je tiens à souligner : la volonté de mettre fin aux retards systématiques du Gouvernement concernant la publication des avis du comité scientifique. Nous sommes ici, je crois, tous d'accord pour dire que la forme de rétention d'informations à laquelle nous faisons face est une anomalie. D'autant que ces avis sont des outils majeurs pour nous permettre d'exercer notre contrôle parlementaire et de légiférer convenablement. Sur l'article 2 encore, je dirai un mot de l'application StopCovid, dont l'utilisation est, hélas, plus que limitée.

Enfin, nous validons pleinement les mesures permettant la réunion des organes délibérants des exécutifs locaux. Si la période est difficile, la vie démocratique est un impératif qui doit aussi suivre son cours. de conserver l'idée selon laquelle un simple avis du préfet est nécessaire pour modifier le lieu de la réunion de l'organe délibérant. Que ce soit dans nos agglomérations, nos territoires ruraux ou encore nos collectivités d'outre-mer, les restrictions sont de plus en plus pénibles pour la population. À nous de continuer le travail de pédagogie auprès de nos concitoyens. En conclusion, je dirai que, vous vous en doutez, mes chers collègues, nous ne votons pas ces mesures de gaieté de coeur, mais l'accélération rapide de la circulation du virus ne nous laisse pas d'autre choix. Vous l'aurez compris, le groupe RDSE votera cette prorogation de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. La parole

pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement nous demandait initialement de proroger le régime transitoire organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 9 juillet 2020, jusqu'au 1 avril 2021. Ce délai a été ramené au 31 janvier par notre commission des lois, afin de permettre une intervention plus régulière du Parlement, ce qui à nos yeux est plutôt salutaire, ne serait-ce que d'un point de vue démocratique. Nous toutefois que le virus circule encore et qu'il circule vite, trop vite. D'autres amendements du rapporteur, Philippe Bas, ont également permis d'améliorer ce texte dans le souci du bon fonctionnement de notre démocratie et de ses instances délibérantes, notamment au niveau local. aucune amélioration n'est selon nous suffisante, comparée au nouveau blanc-seing qui nous est demandé pour attribuer de larges pouvoirs au Gouvernement et aux préfets, pendant plusieurs mois.

Nous ne doutons en rien du constat dressé et de la nécessité des réponses à apporter. Mais une question se pose : ces dites mesures sanitaires adaptées ne sont-elles pas d'ores et déjà à la portée du Gouvernement dans le cadre de notre droit commun ? La réponse est pour nous claire : elles le sont. En cas de recrudescence de l'épidémie, plusieurs dispositifs juridiques pourraient être utilisés. Aussi ce texte est-il, selon nous, aussi dangereux qu'inutile. D'abord, la législation prévoit des dispositions permettant au ministre de la santé de prendre des mesures préventives en cas de danger sanitaire, et la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a spécifiquement prévu le cas de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Ensuite, en cas de nouveau pic de contamination, rien n'empêcherait le Gouvernement de recourir une nouvelle fois à l'état d'urgence sanitaire, par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la santé, comme cela est prévu à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique. J'entends les arguments, notamment de M. le rapporteur, relatifs à ces articles du code de la santé publique. Peut-être faut-il revisiter ces mesures. Mais une chose est avérée aujourd'hui elles sont inscrites dans le code de la santé publique et le Gouvernement aurait pu les dégainer. Enfin, les autorités locales de police administrative- maires et préfets -sont habilitées à adopter toutes les dispositions préventives nécessitées par les circonstances sanitaires locales particulières. En séance, lors de l'examen du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, en juin dernier, nous alertions déjà sur le risque que certaines mesures dérogatoires soient finalement intégrées au droit commun, comme cela s'est produit avec la banalisation des mesures de l'état d'urgence sanitaire pérennisées par la loi dont nous reparlerons demain. Or, précisément, le Gouvernement nous annonce un projet de loi à venir d'ici à janvier 2021, visant à instituer un dispositif pérenne de gestion de l'urgence sanitaire, afin d'éviter « les rendez-vous intermédiaires de prorogation des mesures transitoires ». Le risque est donc bien avéré. Cette loi a créé un nouveau régime juridique, un régime de sortie dans lequel le Premier ministre conserve des pouvoirs exorbitants, notamment celui de réglementer la circulation des personnes, les conditions d'ouverture des établissements recevant du public, ou encore les manifestations et rassemblements sur la voie publique, et celui d'exiger des personnes circulant par voie aérienne sur le territoire national qu'elles présentent un certificat de biologie médicale. Aussi, comme le relève à raison la professeure de droit, Stéphanie Hennette-Vauchez : « [La loi] réduit la voilure de l'état d'urgence sanitaire tel que défini par la loi du 23 mars 2020, mais ce sont bien des pouvoirs exceptionnels de restriction des libertés fondamentales qui demeurent à la main du Gouvernement. » De même, un groupe d'associations, de syndicats, d'universitaires et d'avocats, membre du Réseau de veille sur l'état d'urgence sanitaire, souligne très justement : « Une sortie d'état d'urgence ne s'organise pas, ne s'aménage pas, ne se décline pas : il se lève dans sa totalité pour mettre fin à l'exception. Ce brouillage inédit des frontières est inacceptable. L'exception doit demeurer l'exception et le droit commun la règle. » Alors que le Gouvernement reconnaît que les conditions d'un état d'urgence sanitaire ne sont plus réunies, il estime en même temps nécessaire de maintenir des pouvoirs exorbitants aux autorités administratives. Cette contradiction ne résiste à aucune logique. Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel, indique : « L'état d'urgence ne trouve de justification que dans la faculté pour le Gouvernement de réprimer les manifestations, de limiter les libertés de réunion et les libertés de manifestation. » En effet, à l'heure où les plans sociaux se multiplient, la possibilité accordée au Premier ministre d'interdire les manifestations ne peut que susciter une inquiétude sérieuse. Des pseudo-motifs de santé publique aux véritables raisons politiques, toute la nuance semble se trouver dans ce énième texte d'exception, auquel nous nous opposons.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation sanitaire dans notre pays est grave et s'aggrave. Nous sommes réunis pour la quatrième fois en huit mois afin d'étudier un texte d'exception ayant pour but d'adapter le droit existant à la crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. La situation est grave pour notre santé, mais ce type de projet de loi pourrait être également très grave pour nos libertés

Il y a toujours un risque à vivre libre. C'est à la représentation nationale d'en mesurer le prix et de définir l'éventuel périmètre de restriction que nous serions durablement prêts à consentir. Cela ne peut se faire par voie d'ordonnance ou de décret. Or ce projet de loi permet au Gouvernement, jusqu'au 1 avril 2021, de poursuivre la prise de décret dans de nombreux domaines. Il prolonge également le régime du système d'information de cas contacts covid jusqu'au 1 avril 2021, soit cinq mois, alors que le premier texte, celui de juillet dernier, prévoyait une période transitoire de trois mois et demi. cette durée est inappropriée. Inappropriée en raison de la nature des mesures dérogatoires qui peuvent être prises. Inappropriée parce qu'elle exclut durablement le Parlement d'un débat nécessaire au sein d'une démocratie. C'est pourquoi nous sommes favorables à la proposition de notre rapporteur, votée par la commission, de raccourcir cette durée à trois mois. Ainsi, ce régime d'exception prendra fin en janvier ou, à tout le moins, ne pourra être prolongé sans débat.

Dans le pire des cas, nous prorogerons le délai en connaissance de cause et en fonction de l'inscription de ce projet de loi. À propos de droit commun, je je salue l'initiative de notre rapporteur visant à réécrire l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, ce qui permet de préciser le champ d'intervention du ministre de la santé en cas d'état d'urgence sanitaire. Cette proposition vient consolider juridiquement ce régime de droit commun, qui était à la limite de la constitutionnalité et dont la situation sanitaire actuelle nous a montré l'utilité. néanmoins des points positifs ! Je voudrais particulièrement souligner les apports de nos collègues de l'Assemblée nationale concernant les collectivités locales la possibilité de réunir le conseil en dehors du lieu habituel, la limitation de l'accès au public, ainsi que les visioconférences, sont autant d'outils utiles pour garantir, à la fois, le respect des gestes barrières et la continuité de la démocratie locale. il est préférable pour une collectivité de choisir le meilleur lieu afin de maintenir la tenue de son assemblée, gage de bon fonctionnement démocratique, tout en préservant la santé de ses conseillers.

permettent de concilier l'intérêt médical de cet outil et le respect de la vie privée, qui ne doit pas être oublié, même en temps de crise. Nous avons ainsi voté la « pseudonymisation » des coordonnées électroniques et téléphoniques, comme l'avait préconisé le Conseil constitutionnel le 11 mai dernier, que l'obligation de préciser, dans les décrets qui tendent à créer ces fichiers, une liste limitative de données pouvant être collectées, comme le recommande la CNIL. Je voudrais enfin aborder un point qui n'a malheureusement pas pu être traité dans ce texte par voie d'amendement,

Malheureusement, les études en cours ont été interrompues par le confinement, et 520 POS n'auront pas « fait la bascule » dans les temps. Ce sujet- je viens de le dire -ne pouvant être traité ici et maintenant, je remercie Françoise Gatel de la proposition de loi qu'elle a déposée à ce sujet.

Je pense aussi aux modalités de vote : comment imaginer ne plus voter parce que la covid a encore cours ? Combien de temps nous priverions-nous de vote ? En conclusion, le groupe Union Centriste souhaite revenir rapidement à un État de droit sans exception et, dans sa majorité, il valide cet effort de trois mois encore. Nous voterons donc le texte issu de la commission des lois du Sénat.

que faisons-nous ici, ce soir ? Nous sommes réunis pour la quatrième fois et l'on nous demande de débattre et de délibérer sur la prorogation de l'organisation de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Pour autant, nous ne savons plus très bien de quoi il s'agit. Nous découvrons à l'instant que le Gouvernement a déposé il y a quelques minutes un amendement supplémentaire visant à prolonger des ordonnances prises antérieurement.

été depuis le début- vous le savez, monsieur le ministre -au rendez-vous de la responsabilité. Nous avons travaillé dans des conditions souvent difficiles. Malgré nous ne savons pas très bien quel rôle vous voulez nous faire jouer. Demain- le président de mon groupe l'a rappelé -, le Président de la République s'exprimera ; demain, les grandes chaînes de télévision seront mobilisées.

très attaché aux libertés publiques et au débat parlementaire. Mais nous débattons d'autre chose que de ce qui aurait dû nous occuper, du sujet dont nous devrions être saisis : les mesures privatives de liberté que le Président de la République entend annoncer et imposer au pays. au pays. Pourtant, monsieur le ministre- cela vous a été rappelé tant par le rapporteur que par Mme Assassi à l'instant et par d'autres collègues -, ces mesures sont déjà à votre disposition. En effet, le code de la santé publique est extrêmement bien fait

de détention. Nous le savons- nous sommes tous ici masqués -, le port du masque est obligatoire dans la rue, dans les endroits publics clos, sur les lieux de travail, mais pas en prison.

Le rapporteur, le président Bas, a sans doute voulu préserver la modestie bien connue des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'état d'urgence voté par le Parlement a entraîné une restriction jamais vue de nos libertés publiques et individuelles. Les Français ont accepté d'être mis en quarantaine, d'être « trackés » par une application gouvernementale, de voir leur entreprise couler, d'être mis au chômage, de porter partout et tout le temps un masque, pour la santé de tous. L'état d'urgence est un droit d'exception. Votre régime transitoire est un état d'urgence déguisé. Personne n'est dupe ! Aussi, comme j'avais refusé la prolongation des restrictions de libertés jusqu'au 30 octobre, je la refuse encore plus fortement jusqu'au 1 avril prochain. Le coup de force doit cesser Pour la part qui m'incombe directement, je le dis solennellement ici : les hôpitaux à Marseille n'ont jamais été saturés. Pourtant, hier, sur vos instructions, monsieur le ministre, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de garder les bars fermés deux semaines de plus à Aix-en-Provence et à Marseille. Depuis mars dernier, le ministre de la santé n'a rien fait pour les hôpitaux ni même pour les soignants. Des lits, des postes, du matériel ? Rien ! Aucun investissement immédiat, qui s'imposait pourtant, n'a été consenti. Aucun enseignement n'a été tiré de la première vague de covid de mars dernier. Le ministre de « la santé » porte bien mal son nom : il est en réalité le ministre du confinement et de la restriction des libertés, de la fermeture des bars et des restaurants, de la destruction de la restauration et des centaines de milliers d'emplois de cette filière. vous avez fait fermer les restaurants marseillais et aixois pour quinze jours, avant de les rouvrir sept jours plus tard. Peut-être que, demain, le Président de la République, davantage en père Fouettard qu'en père de la Nation, annoncera de nouvelles fermetures, de nouveaux interdits et de nouvelles restrictions de nos libertés. Plus personne n'y comprend rien, plus personne ne croit en vous, ni même en votre capacité à décider. Vous imposez, vous décidez seul, enfermé dans votre tour d'ivoire, sans jamais consulter les élus locaux et les entrepreneurs. Ne vous étonnez pas, monsieur le ministre, que certains se rebellent contre vos décisions iniques ! Nous traversons une période historique, et vous allez marquer l'histoire : vous êtes sans doute le plus incohérent et irresponsable ministre de la santé de la V République. Pourtant, vous aviez de sérieux concurrents ... La relance économique passera non pas par les ordonnances et les interdits à tout-va, par le retour à l'état de droit et des résolutions garantissant les libertés individuelles et économiques. Pour qu'il y ait relance, il faut qu'il y ait de la confiance. Or, comme des millions de Français, je ne vous fais plus confiance, monsieur le ministre

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis maintenant de nombreux mois, nous sommes confrontés à une situation inédite et anxiogène, à la fois parce que les informations sont souvent contradictoires parce que des dizaines de milliers de nos concitoyens ont été touchés ou le sont encore, tandis que plus de 32 000 personnes sont décédées. Malheureusement, le virus est toujours présent, comme en témoignent les indicateurs de suivi épidémiologique, qui ne sont pas bons dans de nombreux territoires. Cette épidémie n'est pas derrière nous. Le virus circule toujours, parfois de manière très active. Entre le début du mois de juillet et la fin du mois d'août, le nombre des hospitalisations liées au coronavirus et le nombre des personnes en réanimation à cause de la covid ont plus que doublé. La loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire a instauré un régime transitoire, applicable jusqu'au 30 octobre prochain. Ce changement de régime juridique a permis de poursuivre la reprise des activités et le rétablissement du droit commun, tout en conservant la faculté de prescrire des mesures visant à prévenir et, le cas échéant, à maîtriser au mieux une dégradation de la situation sanitaire. Néanmoins, la reprise généralisée des activités amplifie la recrudescence des cas d'infection au covid-19, et cela risque de se poursuivre dans les prochaines Dans ces conditions, une interruption soudaine des mesures sanitaires au 30 octobre ferait courir le risque de laisser se reproduire la catastrophe sanitaire que nous avons connue en mars dernier et qui a contraint à instituer l'état d'urgence sanitaire. Le Gouvernement estime indispensable de conserver, dans les prochains mois, des facultés d'intervention suffisantes pour assurer la continuité de la gestion de crise et prévenir une dégradation de la situation. Dans son avis du 12 septembre dernier, et au regard de l'évolution actuelle et prévisible de l'épidémie au cours des prochains mois, le conseil scientifique a également jugé indispensable de proroger le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire pour une période de cinq mois. À cette fin, le projet de loi initial prévoit de proroger la période de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1 avril 2021. je me félicite de ce que, lors de l'examen en commission, cette date ait été considérée trop lointaine et que la commission ait ramené la durée de prolongation de cinq à trois mois. En effet, compte tenu tant de la nature et de l'intensité des mesures de restrictions susceptibles d'être prescrites que de l'évolution rapide de la situation sanitaire, l'intervention régulière du législateur s'impose, afin de lui permettre de s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité des prérogatives confiées à l'exécutif. Prendre garde à trouver un juste équilibre entre restriction et protection de nos libertés, entre protection de nos concitoyens et protection de nos libertés publiques et de nos valeurs républicaines, apparaît primordial Avant de conclure, je voudrais à cette tribune avoir une pensée pour les nombreuses familles qui ont connu un deuil ou qui, en ce moment même, s'inquiètent pour l'un des leurs. Je pense aussi à tous les soignants et aux personnels de toutes catégories qui sont en première, en deuxième ou en troisième ligne, qui l'ont été, qui le sont de nouveau et qui, hélas, le seront encore si nous ne faisons rien. Monsieur le ministre, mes chers collègues, soucieux de concilier la nécessité de faire face à la pandémie qui nous frappe et le respect des libertés individuelles et publiques, le groupe Les Indépendants et enrichi en commission.

dont l'intitulé comprend des termes devenus éminemment et tristement familiers, y compris pour les nouveaux collègues qui nous ont rejoints il y a peu, et que je salue. En effet, il est question du régime transitoire de sortie de l'urgence sanitaire et, par son biais, de la réponse publique à l'épidémie. Ce régime transitoire, qui prenait la succession de la période si particulière de l'état d'urgence sanitaire, nous en avions discuté aux mois de juin et de juillet dernier. Nous n'avions à l'époque pas obtenu d'accord avec l'Assemblée nationale, alors que nous ne rejetions pas l'idée même d'un régime transitoire. En effet, il s'agit d'un dispositif dérogatoire du droit commun dans lequel le pouvoir exécutif conserve des prérogatives substantielles de nature à limiter certaines libertés. Au regard de la situation sanitaire en juin et juillet derniers, alors en nette amélioration, l'ampleur des prérogatives dérogatoires ne nous avait pas semblé de nature à effectuer le bon arbitrage entre les exigences parfois contradictoires que sont l'impératif de protection de la santé publique et la garantie des libertés individuelles. Cependant, nous avons malheureusement assisté depuis la fin de l'été à une dégradation plus ou moins continue de la situation sanitaire et à un rebond de l'épidémie de coronavirus. Signe de ce regain, 74 départements ont été placés sur la liste des zones de circulation active du virus. C'est dans ces conditions que le Gouvernement a demandé à la représentation nationale de voter la prorogation jusqu'au 1 avril 2021 du régime transitoire, afin de pouvoir poursuivre la mise en oeuvre des mesures et restrictions actuelles. Dans la foulée de cet allongement, l'exécutif a également sollicité une prolongation identique des dispositions créant le fameux système d'information dédié à la lutte contre le covid-19. Notre commission s'est immédiatement saisie du sujet dès le commencement de ses travaux, et a reconnu les nécessités liées à l'évolution de la situation sanitaire. Dans ces conditions, le régime transitoire semble plus à même de concilier les exigences de la santé publique et des libertés individuelles. Nous avons donc souscrit au principe de sa prorogation et de celle du système d'information, mais avec quelques ajustements. Comme le rapporteur a pu le souligner, notre position a été différente sur la durée à donner de cette prorogation. Le Gouvernement suggérait que celle-ci aille jusqu'au 1 avril 2021, soit un allongement de près de cinq mois du dispositif. Cette mesure simplifierait certes la vie de l'exécutif, mais elle serait également de nature à limiter l'intervention régulière du législateur. Or, quand il est question de libertés publiques, de données médicales et de la politique de la Nation face au péril de cette épidémie, nous considérons que faire l'économie de l'intervention de la représentation nationale n'est pas souhaitable. C'est donc à juste titre que notre rapporteur, le président Bas, a proposé de ramener à trois mois ce prolongement, qui durerait donc jusqu'au 31 janvier prochain. Cette position est d'ailleurs proche de celle exprimée par nos collègues députés du En plus de ce choix raisonnable, le texte voté par la commission comprend aussi des aménagements et des améliorations des autres dispositions du projet de loi. Ainsi, nous ne pouvons que nous montrer sensibles à la volonté de prolonger les dispositifs permettant d'adapter le fonctionnement des collectivités territoriales à cette période difficile. Nos élus locaux ont montré tout au long de la crise leur réactivité, leur disponibilité et leur inventivité : il faut continuer à leur faire confiance. Faisons donc le pari de la souplesse à leur égard.

ou encore la reprise des préconisations de la CNIL concernant la fixation d'une liste limitative des types de données pouvant être collectées à des fins de recherche épidémiologique. Enfin, le texte de la commission contient aussi un ajout significatif, qui reprend à l'identique une mesure déjà votée par le Sénat durant son examen de la loi du 9 juillet 2020. Il s'agit de la clarification du régime de droit commun de la réponse aux situations sanitaires graves de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Ces dispositions demeurent trop vagues dans le texte actuel de la loi, ce qui requiert une consolidation, comme l'a d'ailleurs justement identifié le Conseil d'État. Nous espérons que la nouvelle rédaction pourra cette fois Face au rebond de l'épidémie, le texte ainsi amendé offre un équilibre plus satisfaisant, qui, je l'espère, pourra être conservé en commission mixte paritaire. Il est peut-être malheureux que le régime transitoire dure plus longtemps que l'état d'urgence sanitaire proprement dit, mais les outils qu'il offre, ainsi aménagés, semblent appropriés aux exigences de l'heure. Pour ces raisons, le groupe Les Républicains votera le projet de loi dans sa version modifiée. La parole

de la commission ? La commission est défavorable à ces trois amendements, pour la simple raison qu'elle souhaite que le régime issu de la loi dite « de sortie de l'état d'urgence » soit prolongé, et ce pour trois mois.

que nous n'examinerons pas avec beaucoup d'attention le texte en question, que vous n'avez pas encore préparé et dont nous ne connaissons pas le contenu ; je suppose du reste que vous ne le connaissez pas non plus, sans quoi vous nous en auriez parlé

nous souhaitons que soit supprimée la possibilité, pour le Premier ministre, d'interdire la circulation des personnes et des véhicules, tout en conservant la possibilité d'une réglementation. C'est bien l'état d'esprit d'une sortie de l'état d'urgence sanitaire.

de la part des autorités sanitaires. Si des mesures prises étaient jugées disproportionnées par la juridiction administrative, elles seraient bien évidemment annulées. Bien sûr, le Gouvernement aura, si cet amendement est rejeté, un

Le dépôt de plusieurs amendements à ce sujet montre que le sujet est important. Interdire n'est pas justifié dans l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui- ou alors passons directement à l'état d'urgence sanitaire.

Bien qu'ils aient proposé un protocole sanitaire contraignant, ces établissements n'ont pas été autorisés à rouvrir. Il faut aujourd'hui leur permettre de reprendre une activité économique en toute sécurité. Le présent amendement tend donc à proposer que les ERP faisant toujours l'objet d'une fermeture administrative en raison de leur catégorie, parce que leur activité ne pourrait « garantir la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus puissent, sur leur demande, y substituer d'autres activités, proposées par des catégories proches d'ERP et dans le respect d'un protocole sanitaire jugé suffisant par l'administration. Dans une telle hypothèse, les gérants devraient demander au préfet de département l'autorisation de substituer provisoirement à leur activité initiale une activité relevant d'une autre catégorie d'ERP, sans perdre le bénéfice de leur autorisation initiale. Une salle de danse pourrait ainsi envisager de se reconvertir en bar, restaurant, location de salle ou encore salle d'exposition, le temps de sa fermeture administrative.

mais celui-ci n'a jamais été examiné., les activités qu'ils proposent habituellement, en leurs murs, avec professionnalisme, s'exercent- on l'a bien vu, en particulier cet été -de manière sauvage, dans la nature, en dehors de tout encadrement professionnel, ce qui participe pleinement

de sport. En effet, il paraît important que les salles de sport et les équipements sportifs puissent, dans certains cas, rouvrir. Les exploitants de ces salles ont énormément travaillé sur des protocoles sanitaires drastiques, validés par le ministère de la santé,

Par ailleurs, force est de constater que, sur certains territoires, nous arrivons à des situations ubuesques. Par exemple, les salles de sport et autres équipements sportifs de plusieurs métropoles sont fermés,

disposant de prescriptions médicales de sport ne sont plus en mesure d'accéder à leurs soins. Cela peut avoir d'importantes répercussions sur la santé de ces patients. Plusieurs associations se sont élevées contre cette situation.

vise à supprimer complètement la possibilité, pour les autorités sanitaires, de procéder à la fermeture de certaines catégories d'établissements. Il est vrai que, au mois de juillet dernier, nous nous étions opposés à cette disposition, qui figurait dans la loi que nous n'avions pas adoptée.

simple : les restaurants doivent respecter un certain nombre de réglementations- la sécurité incendie, le renouvellement de l'air, etc. Par conséquent, ne devient pas restaurant, même temporairement, qui veut.

promiscuité pouvant présenter un risque sanitaire. Il faut savoir ce que nous préférons ! Le traitement de toutes les difficultés économiques provoquées par les mesures qui restreignent l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie l'industrie doit se faire au travers des mesures de prêt gratuit ou de suppressions de charges, qui sont absolument indispensables pour passer

demandons au préfet de prendre les dispositions pour contrôler la situation. Or, je puis vous l'affirmer, les professionnels qui tiennent ces salles de sport et les collectivités qui ont la responsabilité des équipements sportifs, gymnases et piscines ont pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir correctement le public. Encore une fois, ce n'est pas qu'un problème économique ; c'est aussi un problème de santé publique. Les Français sont encouragés à pratiquer les activités physiques et sportives pour avoir une bonne santé

Je souhaite réagir aux propos de notre rapporteur. Il s'agit de sauver des entreprises qui sont indispensables dans les grandes métropoles, mais aussi dans les stations balnéaires et les communes touristiques, avec des professionnels qui encadrent

de voir des concentrations de jeunes dans des restaurants et de ne pas pouvoir faire la même chose. Aussi, ce qui est demandé ici, c'est que, au cas par cas, le préfet puisse autoriser des activités comparables à d'autres activités de proximité

Ira-t-il jusqu'à les empêcher de vivre pour mieux les protéger d'eux-mêmes ? Le plus grand soin d'un bon gouvernement devrait être d'habituer peu à peu les peuples à se passer lui. » Cette citation n'est pas de moi, elle est de Tocqueville. Ah ! Or j'ai véritablement l'impression qu'elle s'applique aujourd'hui comme en 1838.

leur proposer un changement de catégorie d'ERP, les faire migrer de leur activité, qui subit une fermeture administrative, vers une activité qui fonctionne, fondement d'une décision préfectorale, ne devrait pas poser de problème particulier, puisqu'ils resteraient dans le cadre de la réglementation qui s'applique aux autres ERP. Tel est le sens de mon amendement, auquel il faut répondre plus favorablement

Esther Benbassa. Depuis le début de l'épidémie, en mars dernier, nous n'avons eu de cesse que de dénoncer l'attitude du Gouvernement à l'égard du Parlement. Légiférant systématiquement selon la procédure accélérée, par décrets et par ordonnances, l'exécutif ne laisse que peu de place au législateur dans la gestion de la crise sanitaire. Souhaitant agir avec célérité, il balaie toute velléité de concertation parlementaire, faisant du débat démocratique une variable d'ajustement. Combien de temps encore écartera-t-on les élus des territoires des décisions prises afin d'endiguer la circulation du virus ? Alors que les foyers épidémiques apparaissent localement, il est primordial que les représentants de la Nation et des territoires, députés comme sénateurs, soient davantage informés des évolutions de la pandémie et des moyens financiers, juridiques et sociaux mis en oeuvre pour la

après promulgation de la loi, les discothèques pourraient rouvrir à Paris, à Lille, à Saint-Étienne, à Grenoble, à Marseille, à Aix-en-Provence et dans l'ensemble des zones d'alerte maximale de notre territoire, jusqu'à ce qu'il soit démontré, individuellement, ERP par ERP, discothèque par discothèque, que des foyers identifiés dans ces établissements justifient leur fermeture pour raisons sanitaires. J'indique cela, mesdames, messieurs les sénateurs, parce que j'entends souvent que le Gouvernement est irresponsable, qu'il n'est pas « à la hauteur », pas bon dans sa gestion de la lutte virale. Je veux juste signaler que, avec ce vote, s'il était

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez voté une disposition qui interdit d'office et d'emblée la fermeture d'un ensemble d'établissements recevant du public par catégorie ! Si elle devait être appliquée, empêcherait à tout moment de fermer une catégorie d'établissements, quelles que soient les conditions sanitaires, y compris dans les zones d'alerte maximale. Ne resterait alors que la possibilité pour un préfet de constater qu'un établissement en particulier

la faculté pour les autorités sanitaires de fermer des établissements recevant du public. Est-ce ce que vous avez souhaité en votant cet amendement ? Ou avez-vous pensé que cette disposition allait dans le même sens que les amendements que vous défendiez ?

il serait bon également que le Gouvernement accompagne la caisse des Français de l'étranger dans sa capacité à soutenir ses adhérents qui ne peuvent pas payer leurs cotisations actuellement, compte tenu de l'arrêt ou de la réduction de leur activité, donc de leurs revenus. De nombreux Français vivant à l'étranger ne sont plus en mesure de payer leur assurance maladie en France.

afin de ralentir la circulation du covid-19 au sein de notre population. Le port du masque a d'ailleurs été rendu obligatoire dans certaines municipalités où les contaminations vont et où les hôpitaux commencent à être submergés. Afin de faire respecter cette exigence dans les territoires concernés, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures coercitives afin de responsabiliser nos concitoyens. Désormais, ceux qui se refusent à porter le masque dans les lieux où c'est obligatoire sont susceptibles d'écoper d'une amende, dont le montant équivaut à 135 euros. Le port du masque étant une nécessité de santé publique, nous comprenons parfaitement qu'un dispositif contraignant soit de mise, mais il va sans dire que celui-ci devrait immanquablement être accompagné de mesures sociales, comme la gratuité des masques. Le coût de ces derniers peut en effet devenir un véritable poids financier pour les foyers les plus précaires. À raison de deux masques jetables par jour minimum, la note pour une famille française peut aisément s'élever à plus d'une centaine d'euros par mois. Comment accepter que, en ces temps de crise, de tels frais doivent être assumés par le contribuable, et non par l'État ? Comment accepter que nos concitoyens au RSA, les familles monoparentales, les travailleurs soumis au chômage partiel en raison de la crise économique aient à payer de leur poche le masque rendu obligatoire par les pouvoirs publics ? Ainsi souhaitons-nous qu'un rapport soit remis au Parlement, afin d'évaluer le coût pour l'État que représenterait la gratuité des masques. Il est important que cette information soit communiquée aux parlementaires

C'est un grand classique de nos débats parlementaires, mais il se trouve que ces injonctions au Gouvernement ont un effet nul, d'une part, parce que le Gouvernement n'est jamais obligé de produire les rapports que le législateur exige de lui- la Constitution ne le lui impose d'autre part, parce qu'il ne se prive pas de laisser sans suite toutes ces dispositions quand elles sont adoptées. On se donne bonne conscience à bon compte. Chère

La situation sanitaire justifie de prendre des mesures de police sanitaire, dont certaines affectent directement l'activité de nombreuses entreprises. Dans ce contexte, le présent amendement vise à prévoir des dispositions protégeant les locataires, tout en préservant les intérêts des bailleurs. Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la fin de mesures de police sanitaire restreignant leur activité professionnelle, il est ainsi prévu de faire obstacle aux intérêts et pénalités financières dus pour retard ou non-paiement de loyers ou charges locatives, à la mise en oeuvre des sanctions de l'inexécution ou de l'exécution tardive prévues au contrat, à l'engagement par le bailleur de voies d'exécution forcée, à la mise en oeuvre des sûretés réelles ou personnelles garantissant le paiement des loyers, à la mise en oeuvre de mesures conservatoires. À l'issue du délai de deux mois précédemment mentionné, les bailleurs pourront de nouveau faire valoir leurs droits.

les difficultés que pourrait rencontrer le propriétaire du fait du non-paiement du loyer. Par conséquent, nous souhaitons limiter l'application du dispositif aux seuls loyers et charges locatives concernant les locaux où l'activité de l'entreprise est affectée, et non à d'autres locaux

pour que, en cas de cessation de paiements, le propriétaire devienne un créancier privilégié et puisse entrer ou espérer entrer dans tout ou partie de ces fonds. Tel est l'objet de ce sous-amendement. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ? est favorable au sous-amendement n° 46, qui vise à limiter le périmètre du dispositif aux loyers et charges locatives des locaux où l'activité des entreprises a été affectée par les mesures de police sanitaire.

que les entreprises qui se retrouveraient en difficulté pendant cette période ne puissent faire l'objet de pénalités financières ou d'actions judiciaires de la part de leurs bailleurs en cas de retard de paiement du loyer. L'adoption du sous-amendement contreviendrait à cet objectif, en introduisant une exception consistant à saisir le juge pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires. souligner trois points : l'amendement vise déjà à prendre en compte les intérêts du bailleur ; l'engagement d'actions judiciaires pendant les mesures de restriction de l'activité professionnelle est de nature à créer une relation conflictuelle entre bailleurs et locataires ; enfin, toutes les entreprises ne seront pas concernées par le dispositif : un certain niveau de pertes de chiffre d'affaires

Pourquoi les États-Unis et pas le Canada ? Pourquoi le Panama et pas le Mexique ? Pourquoi les Émirats ou Bahreïn et pas le Qatar ou le Koweït ? ... Personne ne comprend. Les témoignages de nombreux conseillers des Français de l'étranger, aux États-Unis, à l'exemple de celui de Stéphanie Kamaruzzaman, élue de Washington, montrent que l'obtention de ce test préalablement à l'embarquement est parfois impossible dans de nombreux États des États-Unis. Vendredi dernier, l'Assemblée des Français de l'étranger a voté une résolution au nom de l'équité entre ces derniers : elle demande qu'aucune différence ne soit faite entre les Français en provenance des pays listés rouges et que tous puissent passer le test PCR à leur arrivée en France.

Cette situation, qui a fait l'objet d'une ordonnance du Conseil d'État, doit être rectifiée par la loi. En effet, telles qu'elles sont présentées dans le présent projet de loi, les conditions de mise en place des tests de détection dans le cadre des déplacements par transports publics aériens à destination du territoire métropolitain n'offrent pas toutes les garanties constitutionnelles nécessaires. Cet amendement vise à corriger cette situation et à faire respecter le droit constitutionnel au retour sur le territoire national des ressortissants français. L'amendement

les Français et les personnes qui ont le droit de résider en France. Il ne s'agit pas non plus de donner un droit absolu à rentrer sans aucune condition sanitaire.

qui vous invitera à corriger le décret d'application de la loi de juillet 2020, de manière à établir en toute transparence les conditions dans lesquelles vous demanderez aux postes diplomatiques et consulaires de délivrer des laissez-passer sanitaires. Nous ne revenons pas, monsieur le rapporteur, sur l'exigence de sécurité sanitaire, mais nous souhaitons la transparence sur les conditions dans lesquelles les laissez-passer sanitaires seront délivrés. Aujourd'hui, les postes consulaires sont livrés à eux-mêmes, sans instruction transparente,

son statut sérologique étant connu, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se soigner. Il me semble

au retour sur le territoire national ne sont applicables que pour quatre pays de provenance : le Bahreïn, les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Panama.

les frontières sont fermées avec les pays dans lesquels le virus est considéré comme très « circulant ». Seules peuvent donc entrer en France les personnes qui sont résidentes françaises ou de nationalité française ou en situation exceptionnelle. On classe ces pays

Ce qui me paraît important dans ce débat, monsieur le ministre, c'est que vous preniez acte d'un certain nombre de faits qui nous sont rapportés par nos collègues sénateurs représentants des Français de l'étranger. Ces faits sont simples une partie de nos compatriotes, même dans un grand pays comme les États-Unis, n'arrivent pas à obtenir dans un délai suffisamment bref les résultats d'un test. Dès lors, que fait-on pour eux ?

M. Olivier Cadic. Les personnes arrivant en France en provenance d'un pays énuméré dans l'annexe II du décret du 10 juillet 2020 doivent se soumettre à la réalisation d'un test de dépistage virologique à leur arrivée à l'aéroport, à défaut d'avoir pu réaliser un tel examen biologique dans les 72 heures précédant le départ. Il semble toutefois que les tests sont réalisés de façon extrêmement aléatoire, même s'agissant de voyageurs provenant de pays où la situation sanitaire est catastrophique.

aux voix l'article 1A. ter Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 20 amendements au cours de la journée ; il en reste 26 à examiner sur ce texte.